La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 13 février de la suite de la nouvelle lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la nouvelle lecture du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, avant l'examen du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la Polynésie française. En conséquence, le Gouvernement demande également l'inscription à l'ordre du jour du jeudi 14 février, le matin, l'après-midi et, éventuellement, le soir, à l'issue de l'examen de la proposition de loi relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte, de la suite éventuelle de l'examen du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la Polynésie française. Acte est donné de cette demande. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en

qui prévoit que l'entrée en fonction des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection. amendement vise à ce que les sociétés concernées ne soient pas obligées d'organiser une assemblée générale six mois après celle qui aura permis de modifier les statuts. L'organisation de cette nouvelle assemblée générale en cours d'exercice pourrait en effet représenter des coûts importants dans les grandes sociétés.

n° 458 rectifié comporte plusieurs dispositions visant à réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi qu'avait déposée Nicole Bricq en 2008. La plupart des dirigeants de société jouissent d'un contrat de travail « officiellement suspendu »- terme quelque peu ambigu -durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu'ils puissent toucher des indemnités de départ. En raison de ces ambiguïtés, le 1° supprime le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive à seule fin de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail. Dans le même esprit, le 2° supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d'administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d'administration.

sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d'un préjudice, direct ou indirect, qu'ils auront pu personnellement subir. Le II prévoir la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L'irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive ; il convient donc d'obliger le dirigeant comme l'administrateur dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.

La persévérance est une qualité, sauf quand il s'agit de persévérer dans l'erreur, mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Avec cet amendement, nous revenons sur la question de la transparence des rémunérations. La mesure de l'écart des salaires par rapport au salaire moyen ou au salaire médian n'est pas suffisante et ne permettra pas de lutter contre les inégalités salariales.

tend à prévoir un avis conforme du comité d'entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d'administration. Afin d'aider le conseil d'administration à assumer ses choix, le II vise à mettre en place un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d'administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations du président du conseil d'administration. Le III tend à tend à assurer l'information de l'assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.

objet d'instituer un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et

à conditionner les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d'administration et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.

Mais la perception des écarts de richesse est, quant à elle, restée d'ordre national, et nos concitoyens, on le voit actuellement, y sont particulièrement sensibles. En outre, certains pays pratiquent une modération salariale qui ne les empêche nullement d'attirer les talents internationaux. Ainsi, le Japon est, avec le Danemark,

Il est devenu contraignant depuis la loi Sapin II et nous proposons que de telles rémunérations soient soumises également à un avis conforme du comité social et économique, qui a remplacé le comité d'entreprise. Au Danemark, Au Danemark, l'écart entre les plus hauts salaires et le salaire moyen est de 1 à 20, quand, en France, il est de 1 à 77. Nous proposons qu'une limitation identique s'applique dans notre

de le redéfinir, mais en faisant bien la distinction entre ce qui relève du législatif, du respect des règles, et ce qui relève de l'incitation.

pour les rémunérations différées. Au-delà d'un montant de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de société

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 62 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Cet article visait à garantir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions exécutives des sociétés.

respecter la loi. Invoquer un possible contournement de la loi pour s'abstenir de légiférer, c'est ériger le renoncement en méthode de gouvernement. Pourtant, on nous répète à longueur de temps que c'est la « confiance » qui doit présider à nos relations avec les entreprises. Nous proposons donc de rétablir le dispositif de l'article 62 . Pour rappel, l'article 1 de la Constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Cela nous impose de ne pas renoncer au prétexte que quelques entreprises ne seraient pas vertueuses. Il faut au contraire agir en fixant un objectif ambitieux.

Je suis profondément attaché à la parité et la féminisation des fonctions de direction. Je considère que l'entrepreneuriat au féminin- j'ai eu l'occasion de le dire ce matin -est une des clés de la reconquête économique de notre pays. J'ai le sentiment que si on ne met pas un peu plus le pied dans la porte, on n'y arrivera pas.

qui ne respectent pas leurs obligations légales en la matière. À l'heure actuelle, et malgré les lois successives en matière d'égalité professionnelle, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes restent élevés, puisque la différence est de 27,5 %, tous temps de travail confondus.

faut, nous semble-t-il, sanctionner davantage les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. La loi impose aux entreprises, au-delà d'un certain effectif salarié, de négocier un accord d'entreprise ou d'élaborer un plan d'action en matière d'égalité professionnelle. Or 60 % seulement d'entre elles se sont pliées à cette obligation. Des sanctions sont prévues pour les entreprises récalcitrantes. L'inspection du travail peut mettre en demeure une entreprise ayant manqué à ses obligations. Elle peut entendre les justifications du chef d'entreprise et, en dernier recours,

commission spéciale, tendait à prévoir la nullité des délibérations du conseil d'administration en cas de non-respect de la règle imposant la présence 40 % de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Dans la mesure où la règle des 40 % de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance est respectée par une très grande majorité d'entreprises, il ne nous paraît ni disproportionné ni dangereux que

est à Mme Laurence Cohen. L'article 62 vient modifier les règles relatives au droit à l'information préalable des salariés, en créant une obligation d'information des salariés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de leur entreprise, ce qui est une avancée positive.

reprendre l'entreprise. Ensuite, cet article vient restreindre l'obligation faite aux employeurs, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, d'informer au préalable leurs salariés lorsqu'ils envisagent le transfert d'un établissement dans la même Cette obligation se justifie pleinement, car un tel transfert est susceptible d'entraîner des conséquences sur la marche générale de l'entreprise et sur les conditions de travail, donc sur les salariés. Le chapitre III de ce projet de loi est sous-tendu par l'ambition de rendre les entreprises plus justes et de modifier leur place dans la société. Pourtant, l'article 62 s'inscrit dans la droite ligne des réformes précédentes, qui consistent à déresponsabiliser les entreprises en limitant leurs obligations à l'égard des salariés et en privant ceux-ci de la possibilité de prendre part aux décisions relatives à la marche de l'entreprise. Le groupe CRCE avait, lui, pour ambition de renforcer la participation des salariés aux prises de décision dans l'entreprise. C'est pourquoi nous avions présenté une série d'amendements visant à accroître le rôle des salariés et des représentants du personnel, en renforçant leur droit à l'information et en rendant plus effectifs leurs pouvoirs d'intervention. Aucun de ces amendements n'a été jugé comme étant en lien avec ce texte, alors même qu'ils contribuaient à repenser la place de l'entreprise dans la société Hier soir, Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances a pris exemple sur l'Allemagne pour justifier la réduction du taux du forfait social. Il est dommage que le Gouvernement ne s'inspire pas du modèle allemand

vous tentez ici d'abroger ce dispositif, qui se limite pourtant à prévoir une obligation d'information des salariés deux mois avant la vente ou la reprise d'une entreprise. Nous sommes qui concerne toutes les entreprises, est beaucoup plus long. La suppression de cette obligation constituerait une grave erreur. Il est vrai que certaines reprises ne posent aucun problème, mais il arrive que les repreneurs soient des prédateurs ou soient tout simplement « bidons » ! Les salariés, notamment les cadres, sont alors à même de s'en rendre compte.

l'entreprise ne saurait évoquer avec ses salariés les conditions de la reprise deux mois avant la vente, c'est à l'évidence un recul social.

Christine Lavarde. L'exposé des motifs de l'article 62 précisait que le droit d'information préalable était destiné à remédier à la non-transmission d'entreprises saines. Il aurait donc vocation à s'appliquer uniquement lorsqu'il n'y a pas de repreneur. Or le texte va aujourd'hui au-delà,

: La parole est à M. Franck Menonville. Cet amendement concerne le droit d'information préalable des salariés en cas de vente de l'entreprise, qui, malgré des intentions tout à fait louables, suscite parfois

Ce droit serait applicable dans les entreprises employant jusqu'à 249 salariés. Il s'agit de privilégier la reprise de l'entreprise par celles et ceux qui ont à coeur la préservation de l'emploi, de tous les emplois, au contraire des repreneurs qui considèrent systématiquement l'emploi comme une variable d'ajustement et ne cherchent qu'à assurer un taux de profit acceptable pour les actionnaires. C'est un amendement que nous présentons depuis de nombreuses années. À chaque fois, il nous est répondu que ce droit de préemption des salariés ne serait pas constitutionnel eu égard au droit de propriété,

Pourquoi en irait-il autrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou d'une usine ? Il ne s'agit pas de priver qui que ce soit de ce qui lui revient, puisque l'exercice du droit de préemption oblige à racheter l'entreprise au prix légitimement fixé. C'est une proposition d'intérêt général, qui vise à replacer l'emploi au coeur des préoccupations économiques, en s'appuyant sur de nouveaux droits pour les salariés.

anglo-saxon. Il s'agit non pas de reconnaître à ces dernières des droits indus, mais uniquement de prévoir une préférence de rachat en cas de vente ou de transmission.

Ces dispositifs, plus connus sous le nom de retraites « chapeau », permettent à des salariés, généralement très haut placés, de toucher une prime importante, qui s'ajoute à leur pension de retraite légale. Ils ont fait scandale ces dernières années en raison des montants astronomiques en jeu. Par exemple, le montant de la retraite « chapeau » du PDG de GDF Suez avait suscité la polémique il y a quelques années : supérieur à 830 000 euros annuels, il avait de quoi surprendre et choquer, d'autant que GDF Suez avait terminé l'année 2013 sur une perte de près de 10 milliards d'euros Cet article 65 vise à donner la main au Gouvernement pour réformer un dispositif permettant à de hauts cadres, dont les revenus sont déjà très élevés, de toucher des primes faramineuses.

estimé préférable la codification des dispositions relatives aux activités de ces agences dans le livre II du code de commerce au prétexte qu'elles qu'elles s'adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. En réalité, le livre II du code de commerce est exclusivement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités sont toutes traitées dans le code monétaire et financier, à l'image des services bancaires, des services de paiement et des services d'investissement. Ce qui nous intéresse ici, c'est non pas la forme juridique des agences de conseil, mais leur activité. Il s'agit d'un amendement de pure cohérence juridique.

En outre, la commission spéciale a clarifié la rédaction de ces dispositions tout en restant fidèle à la directive concernant l'engagement à long terme des actionnaires, ce que l'amendement ne prend pas en compte.

Yung, pour explication de vote. Je suis évidemment favorable à la transposition de ces directives. Nous menons un combat permanent contre toutes les formes de contrefaçon, et nous avons eu un débat très difficile avec la Commission

relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement. En effet, cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1 janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraîne, de fait, un déséquilibre dans la relation entre le prêteur et l'emprunteur, en défaveur du consommateur.

concernait que deux réseaux bancaires sur six -et qu'il était également très contesté. L'opposition émane des associations de protection des consommateurs, des intermédiaires en crédit et des syndicats représentant les personnels des établissements bancaires.

Je suis favorable à cet amendement, qui tend, d'une part, à apporter des corrections relatives aux modalités de souscription et de rachat de titres de créances, et, d'autre part, à préciser la notion de « sponsor » pour les organismes de titrisation, avec une référence plus pertinente.

dite « DEVF ». Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l'organisateur ou du détaillant d'un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit Ainsi, l'agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage. Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres États membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors que ceux-ci se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne. Les compagnies d'assurances se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d'assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans davantage de garanties pour le consommateur. Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l'organisateur de voyage prévues à l'article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l'article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.

celle-ci, il n'y a pas de définition du régime de responsabilité. Le maintien de la responsabilité de plein droit ne constitue donc pas une sur-transposition.

rien à voir avec les voyagistes ! Il s'agit de ratifier deux ordonnances, sur le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. J'insiste, il s'agit

auprès d'un courtier ou d'une société d'assurance ; or, quand elles souhaitent la faire jouer, la société, qui curieusement est domiciliée à Chypre, Malte ou Gibraltar, a disparu.

Je vous ai expliqué les cas que nous visions. Face à cette situation, il est urgent d'améliorer les conditions de commercialisation des produits d'assurance. C'est dans cette perspective que nous proposons de mettre en place un dispositif d'autorégulation en obligeant les courtiers d'assurances et les IOBSP à adhérer à des associations professionnelles représentatives agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, qui pourra ainsi l'activité de ces courtiers. Ces associations rempliraient des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification, etc. De plus, elles disposeraient d'un pouvoir

un avis défavorable spéciale ? Si l'ordonnance tend au renforcement des pouvoirs de l'instance qui immatricule les courtiers d'assurance, l'impact de cette mesure n'est pas précisé. En outre, nous venons d'adopter à l'instant les amendements identiques de MM. Bizet et Yung sur la nouvelle instance interprofessionnelle qui permettra à l'ACPR d'assurer un meilleur contrôle de ces acteurs.

par ordonnance la directive qui harmonise les prérogatives des autorités nationales de concurrence et, d'autre part, de renforcer l'efficacité des procédures de l'Autorité de la concurrence et des enquêtes de la

Cet amendement vise à insérer un article dans le code de commerce pour encadrer les conditions dans lesquelles les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF ont accès aux données de connexion,

dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l'énergie. Depuis 2002, différents gouvernements ont donné quitusà la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l'énergie. Hier, en 2002 comme je viens de le à la concurrence totale. Aujourd'hui, ce sont les dernières protections que sont les tarifs réglementés pour les consommateurs qui disparaissent. En effet, sont concernés le gaz et l'électricité pour les très grandes entreprises, un prélude à la suppression totale des tarifs réglementés. Cela est inquiétant. De surcroît, on nous demande de légiférer contre ces droits acquis que sont les tarifs réglementés du gaz sans la moindre étude d'impact. On nous dit : « Votez les yeux fermés

Nous avons même déposé par le passé des propositions de loi en ce sens. Cela dit, et compte tenu de la décision du Conseil d'État, nous ne pouvons faire autrement que de nous incliner. En réalité, nous n'avons pas le choix ! C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas déposé d'amendement de suppression de l'article, même si nous en avions fortement envie.

en 2007. L'État ne fixera plus par arrêté les tarifs que doit proposer aux consommateurs l'opérateur historique, pour laisser libre la concurrence entre fournisseurs d'énergie. L'argument est toujours le même : l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel est l'occasion de donner aux entreprises de ce marché de nouvelles occasions de croissance et d'innovation, tout en permettant aux consommateurs de bénéficier d'une fourniture de gaz naturel adaptée à leurs besoins. comment ignorer que, depuis 2007, sur les 10,6 millions de consommateurs abonnés au gaz, 5,4 millions de particuliers et 73 000 professionnels sont encore titulaires d'un contrat au tarif réglementé ? La concurrence par le marché n'a pas fonctionné. Vous organisez donc la concurrence pour le marché ! À cet égard, la cohérence de cette disposition va avec la cession des parts d'Engie. nous pensons que la question des tarifs réglementés de l'énergie exige un débat à part entière. Nous devons prendre le temps ici d'en discuter véritablement, d'autant que- vous le savez fort bien -la fin des tarifs réglementés ne rencontre pas l'assentiment de nos concitoyens. Le tarif réglementé est en effet la garantie d'un tarif qui dépend moins de la fluctuation des marchés financiers. S'il fonctionne aujourd'hui comme un plafond, c'est tant mieux Vous savez aussi fort bien que la fin des tarifs réglementés voulue par la Commission européenne se traduira par une explosion des tarifs du gaz et de l'électricité pour les particuliers. Enfin, monsieur le ministre, nous avons besoin d'un ministre non pas spectateur dans ces négociations, mais acteur. Vous pouvez le faire, comme vous en avez fait la démonstration sur les GAFAM.

mais un certain nombre d'éléments font qu'il me paraît justifié de transposer cette directive, en ménageant une transition qui soit la plus douce possible. La décision du Conseil d'État indique très clairement que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont désormais contraires au droit européen. Si nous ne transposons pas rapidement cette mesure, nous allons exposer des clients

; il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas soumises à une remontée brutale des tarifs ou à des coupures de gaz parce qu'elles ne pourraient pas payer leurs factures. Nous avons pour cela créé un dispositif de fourniture de dernier recours

mais qui doit être plus précis et plus pertinent, afin d'informer les consommateurs. Tel ne nous paraît pas être le cas avec l'amendement présenté par le Gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous n'y sommes pas favorables. Je mets

Mme Jacky Deromedi. Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas nécessairement aux seuls tarifs réglementés, sauf à considérer que la suppression de ces tarifs, au plus tard à compter du 1juillet 2023, mettra fin à toute possibilité d'intervention publique dans le champ de la fourniture de gaz naturel à l'échelon local, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. En effet, comme on a pu s'en rendre compte au cours des derniers mois, nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité. Au demeurant, le présent amendement est cohérent avec les dispositions du III du présent article, qui prévoient de maintenir l'habilitation dont bénéficient les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour exercer des missions de conciliation en vue du règlement de certains différends, en l'occurrence ceux relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121-32 du code de l'énergie. Il est toutefois indispensable de permettre aux autorités précitées de contrôler également la mise en oeuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où cette mission de service public, applicable aux consommateurs résidentiels qui ne parviennent pas à trouver un fournisseur de gaz naturel, est directement liée au thème de la précarité énergétique, et où de nombreuses initiatives concrètes sont prises à l'échelon local, sous la responsabilité aussi bien des autorités chargées de l'action sociale que de celles qui sont également impliquées dans la résorption de ce phénomène, directement ou indirectement, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. de leurs compétences. Quel est l'avis de la commission spéciale ? L'amendement a pour objet que l'activité d'un fournisseur de dernier recours ou de secours soit encadrée par les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel. Bien que je sois attaché au rôle et aux prérogatives de ces autorités, il me semble qu'il ne leur appartient pas de fixer les conditions dans lesquelles la fourniture de dernier recours ou de secours devra s'exercer. Ces conditions seront en effet fixées par les cahiers des charges des appels à candidatures qui seront organisés par le ministère, avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie. Une fois les fournisseurs désignés par zone de desserte,

Cet article, issu de l'adoption en commission spéciale d'un amendement de M. le rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi des dispositions relatives au gaz naturel pour lesquelles l'article 71 dans sa rédaction initiale, habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Nous sommes favorables à cette proposition, qui permet d'éviter le recours aux ordonnances et laisse donc au Parlement la possibilité de se prononcer sur les dispositifs de fourniture de dernier recours et de dernier secours. Nous sommes favorables à de tels dispositifs, dont nous avons réclamé la mise en place depuis longtemps, pour le secteur du gaz naturel comme pour celui de l'électricité. Ces dispositifs sont utiles, même lorsqu'il existe des tarifs réglementés. Plus encore, ils sont particulièrement nécessaires du fait de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel actée par la Commission européenne, validée par le Conseil d'État et à laquelle nous nous sommes toujours opposés. Nous regrettons cependant que le dispositif de fourniture en dernier recours pour les clients ne trouvant pas de fournisseur de gaz naturel en limite le bénéfice aux consommateurs « domestiques » de gaz naturel. En effet, le versement d'un dépôt de garantie peut être exigé par le fournisseur lors de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz naturel. Avec la fin programmée des tarifs de vente de gaz naturel, le risque que certaines entreprises ne puissent souscrire un contrat en raison des exigences du fournisseur en matière de dépôt de garanties est bien réel. Selon le médiateur national de l'énergie, lors de la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité de plus de 36 kVA, des professionnels en difficultés financières n'ont pu souscrire un contrat en raison du montant prohibitif de dépôt de garantie exigé par le fournisseur historique lui-même lors du passage en offre de marché. Face à de tels risques, nous proposons d'élargir le bénéfice du dispositif de dernier recours, en ne le limitant pas aux seuls clients domestiques.

La commission spéciale y est favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 1008, qui a pour objet, par coordination, que le cahier des charges de l'appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours précise, comme c'est déjà prévu pour la fourniture de secours, les catégories de clients couvertes.

l'amendement n° 284 rectifié. La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur. La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés. Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d'électricité ou de gaz, notamment en cas d'impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, laquelle relève plus largement de l'action sociale. Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d'en haut, c'est-à-dire au niveau national.

il s'agit de mettre en place un recueil de l'accord du consommateur au tarif réglementé de vente, pour transmettre ces données au fournisseur qui en ferait la demande : accord exprès jusqu'au 30 septembre 2022, accord tacite ensuite.

Cet amendement tend à préciser certaines des modalités d'information des consommateurs sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz. Il s'agit de donner un délai suffisant aux fournisseurs pour délivrer cette information.

ce qui concrétise l'engagement pris par le Gouvernement dans l'objet de son amendement initial. Au vu du nombre de clients concernés, une communication encore plus large sera certainement souhaitable, mais seul le Gouvernement pourra la prévoir dans la loi, du fait des règles de l'article 40 de la Constitution. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous éclairer sur ses intentions

qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture. Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n'est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Dans ces conditions, il convient de préciser que l'abrogation de cette disposition n'entrera en vigueur que le 1juillet 2023.

Il nous faut donc organiser la sortie progressive des autres clients dans les meilleures conditions. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise quatre grands objectifs. Premièrement, il s'agit de faire jouer au Parlement son rôle plein et entier sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et de fixer des règles claires dès à présent. convient d'assurer la transition la plus progressive possible, en organisant une sortie « en sifflet » selon les catégories de clients concernées et en donnant du temps pour éteindre les contrats en cours d'exécution. il faut clarifier le sort réservé à certains types de clients, en prévoyant que les copropriétés, de même que les petites collectivités territoriales et les petites associations, pourront continuer à bénéficier des tarifs. nécessaire d'assurer la meilleure information et la meilleure protection possible des consommateurs, sur le modèle de ce que nous avons déjà prévu pour le gaz. À ce stade, le Gouvernement n'est pas favorable, si j'en crois l'amendement de rétablissement de l'ordonnance qu'il a déposé par ailleurs, à cette législation directe sur l'électricité. Mais je ne désespère pas de le convaincre du bien-fondé de la démarche d'ici à la commission mixte paritaire, voire, si nous devions échouer en CMP, de persuader nos collègues députés qu'un tel sujet ne peut être traité par ordonnance, sans connaître ni le périmètre précis des clients éligibles

à M. Roland Courteau. Cet article, issu de l'adoption en commission spéciale d'un amendement de M. le rapporteur, vise à introduire dans la loi le dispositif relatif au comparateur d'offres d'électricité et de gaz naturel, sur lequel l'article 71 prévoyait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Nous considérons néanmoins que, pour ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d'application du comparateur à 30 000 kilowattheures n'est pas pertinente. Aujourd'hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu'à 300 000 kilowattheures par an ; elles concernent par exemple des PME ou de petites copropriétés qu'il ne paraît pas légitime d'exclure du dispositif. Nous proposons donc, par cet amendement, de modifier le seuil prévu par cet article, de

n° 484 rectifié . En introduisant dans la loi les dispositions relatives au comparateur d'offres d'électricité et de gaz naturel, M. le rapporteur a prévu qu'un arrêté vienne préciser les modalités d'application du dispositif prévu par l'article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur ». Nous souhaitons supprimer ce renvoi qui ne paraît pas pertinent, pour plusieurs raisons ; en particulier, le statut même du médiateur national de l'énergie, en tant qu'autorité publique indépendante, est une garantie d'objectivité et de non-discrimination à l'égard des fournisseurs. Les informations enregistrées font l'objet d'un encadrement strict qui garantit une présentation des offres transparente, objective et non discriminatoire. Il est donc selon nous inutile de prévoir un tel arrêté ; celui-ci serait non

Ce marché carbone est actuellement considéré comme le principal levier des politiques climatiques européennes, permettant de rendre l'industrie compatible avec une économie bas carbone.

sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. En effet, le relèvement du seuil de contrôle légal et de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes aura, à n'en pas douter, des répercussions importantes et potentiellement déstabilisantes. Les modifications apportées par le Sénat, qui contribuent notamment à améliorer la rédaction de ce dispositif, ne dispensent pas d'une telle évaluation. Un comité d'évaluation composé de parlementaires serait donc constitué au plus tard dans les trois ans après la promulgation de la loi PACTE ; il s'attacherait à réaliser le bilan des effets de l'absence de certification légale sur l'économie française, en matière notamment d'accès des entreprises au financement, de croissance des entreprises, de sécurité financière et de délinquance économique. Le bilan porterait également sur l'évolution du marché de l'audit

tous les sénateurs de la qualité des débats que nous avons menés. Nous n'avons pas été d'accord sur tout, c'est très clair, y compris s'agissant de points fondamentaux de ce projet de loi. Néanmoins, nous avons eu un débat approfondi, à la hauteur des enjeux économiques et démocratiques de ce texte, et je tenais, une fois encore,